monsieur le président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

sur les dix dernières années de libéralisation du secteur de l'énergie. Alors que se sont multipliés les prestataires de fourniture- vingt et un aujourd'hui -et alors que la gestion du réseau de distribution fait toujours l'objet d'un duopole Enedis-GRDF, il est nécessaire de faire un point d'étape. Le premier constat que l'on peut tirer, c'est que l'ouverture à la concurrence a au final peu convaincu, avec 15 % du marché de l'électricité et 25 % de celui du gaz, principalement dans le secteur des entreprises. Mais ces quelques données ne font pas un bilan qualitatif ni sur l'amélioration du service rendu aux usagers ni sur les tarifs pratiqués. Pis, c'est ce qui a finalement ouvert la porte au Conseil d'État, à la suite du recours de pour remettre en cause les tarifs réglementés du gaz. Il est vrai qu'à la différence de l'électricité cette énergie n'est pas considérée comme un produit de première nécessité au sein du code de l'énergie. Toutefois, la mesure ne pouvait que fragiliser la situation économique des plus précaires, car parler d'énergie substituable implique de pouvoir changer soit de raccordement, soit de matériel. La substitution est donc moins automatique qu'il autre motif qui devrait alerter ou du moins conduire à s'interroger est le nombre important de recours déposés devant le Conseil d'État. Dernier élément, la baisse des prix de l'énergie promise est absente, et l'impossible retour aux tarifs réglementés une fois le choix du prix du marché effectué pose question. On se retrouve dans une situation où il est possible de revenir à l'offre publique, mais uniquement au prix du marché. Ainsi, entre 2007 et 2015, la facture d'électricité s'est envolée de 49 % et celle du gaz de 36 %. On parle de presque 2 000 euros par an et par ménage pour une énergie pourtant nécessaire. De fait, cette situation impose aujourd'hui un état des lieux complet des résultats de la libéralisation du secteur, tant quantitativement que qualitativement.

n'est pas favorable à un nouveau rapport. J'invite d'ailleurs notre assemblée à se saisir de toutes les possibilités de contrôle qui sont à sa disposition, car l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même

Mais elle a ajouté : « La situation est plus compliquée sur les marchés de l'énergie. Il faut raisonner marché par marché, sans calquer un modèle unique.

apportées, nous n'avons pas intérêt à voir se réduire la part de l'État et la maîtrise publique au sein d'une entreprise exerçant dans un secteur aussi stratégique que l'énergie. Il y va de notre sécurité d'approvisionnement et de notre souveraineté énergétique que l'État continuera d'édicter la régulation et conservera l'action spécifique lui permettant de s'opposer à toute décision de cession d'infrastructures stratégiques, je persiste à voir dans cette suppression du seuil minimal plusieurs risques pour l'évolution tarifaire supportée

le devenir de certains actifs stratégiques après la privatisation- stockage souterrain de gaz, réseau de transport -dès lors que l'action stratégique relève seulement du pouvoir réglementaire. Par ailleurs, qu'en pensent les salariés, qui ont déjà constaté la destruction d'emplois, alors que l'entreprise délocalise dans des pays à faible coût de main-d'oeuvre ? Qu'en pense également François de Rugy ? Comment pourra-t-on s'assurer que cette entreprise où l'État aura quasiment abandonné sa part continuera d'emprunter le chemin de l'énergie verte et de la transition énergétique et écologique ? Comment le Gouvernement pourra-t-il s'assurer qu'Engie persistera à se positionner

Dans le secteur de l'énergie, la libre concurrence généralisée n'est pas la bonne stratégie ! Deuxièmement, nous avons besoin d'investissements de long terme pour la transition énergétique, en particulier en ce qui

nous permettrait, en tant que parlementaires, d'avoir un regard cohérent dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, de la stratégie nationale bas carbone, des territoires à énergie positive, en liaison bien sûr avec les autorités concédantes, les concessionnaires

non pas d'une entreprise nationale produisant et préservant les sources d'énergie en France, mais, par définition, d'une entreprise tournée vers la compétition internationale qui doit faire face à des entreprises américaines, britanniques, indiennes, lesquelles

encadrer les privatisations et assurer le rôle central de l'État. Il n'avait fallu que deux ans au législateur pour passer d'une entreprise pleinement publique à une société anonyme, sans majorité étatique de contrôle, en passant par une période dite « tampon » pendant laquelle la propriété publique était garantie à 70 % au moins du capital social. Puis 2014 fut l'année de la seconde banderille, avec une distinction entre détention de capital et détention des droits de vote pour affaiblir encore la présence de l'État. Monsieur le ministre, vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous ne comptiez pas refaire les erreurs commises lors des privatisations passées, notamment celles qui découlent de la mise en concession des autoroutes. Nous aurons, d'ici à quelques semaines, l'occasion de revenir sur ce sujet.

Premièrement, nous regrettons que le Gouvernement fasse une nouvelle fois le choix de renoncer à des rentrées d'argent. Monsieur le ministre, on ne peut pas en même temps déplorer le déséquilibre budgétaire de l'État et refuser la part des 350 millions d'euros de dividendes que lui verse Engie chaque année- cela en fait d'ailleurs l'une des trois entreprises qui distribuent

en matière de transition écologique. De fait, la lutte contre le réchauffement climatique et la rationalisation énergétique sont le combat de ce XXI siècle,

ainsi qu'à l'ouverture du capital de GRTgaz. C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de l'article 52. Nous considérons qu'une participation importante de l'État au capital d'une entreprise aussi stratégique constitue

nous continuons à nous inquiéter du devenir de certains actifs stratégiques après la privatisation des réseaux de transport de gaz naturel, mais aussi des actifs de stockages souterrains de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, le GNL, les droits attachés à cette action spécifique relevant du pouvoir réglementaire. Nous estimons par ailleurs que dans le contexte actuel de financiarisation de l'économie, l'État doit rester fortement présent au capital d'Engie, afin d'éviter la captation d'une grande part de la valeur créée au détriment de toutes les parties prenantes et un repli sur des choix de court terme, en particulier en matière d'investissement- optimisation fiscale, rachat d'actions ... -, typiques du capitalisme actionnarial actuel

? Je rappelle aux auteurs de ces amendements qui s'inquiètent du devenir des infrastructures appartenant à Engie et à GRTgaz, et qui souhaitent que l'État garde la maîtrise et le contrôle des entreprises de l'énergie- j'ai même entendu parler d'un pôle public de l'énergie

... Je l'ai déjà dit, le contrôle de la puissance publique continuera à s'exercer par le biais de deux instruments qui sont loin d'être négligeables : d'une part, le secteur restera régulé sous l'égide de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE ; d'autre part, l'État disposera toujours, et cela a été rappelé, d'une action spécifique lui permettant de s'opposer à la vente d'actifs jugés stratégiques.

! Je préfère rester sur du solide. Le solide, c'est ce que nous vous proposons en matière de cession d'actifs depuis hier. En effet, la logique et la cohérence sont les mêmes pour toutes ces opérations

permettre à notre pays de se développer économiquement de manière plus rapide, en investissant dans l'innovation et, en l'espèce, dans les énergies renouvelables. La situation d'Engie a été rappelée par chacun d'entre vous : l'État, qui a un peu moins de 24 % du capital et 34 % des droits de vote, est limité dans ses évolutions par la loi puisqu'il ne peut pas descendre en deçà des 33 % de droits de vote. Si Engie veut se développer,

aux installations de gaz naturel liquéfié. Toutes ces installations sont protégées par l'action spécifique et ne peuvent donc être cédées ni par Engie ni par ses filiales.

la rémunération des dividendes est liée non pas à la baisse de chaque action, car les dividendes ont fortement crû dans 90 % des entreprises, mais à la réduction de la voilure. À force de privatiser, la masse d'actions qui sont rémunérées ne cesse de baisser, et les études sont claires en la matière

S'agissant de l'État stratège, je n'ai aucune difficulté à reconnaître que l'État doit intervenir par moments et investir dans une entreprise qu'il estime stratégique. Prenez l'exemple d'Ascoval.

Qui peut croire aujourd'hui que les entreprises publiques sont les seules garantes d'un service public de qualité ? Il me semble que cet argument est un dogme. Si toutes les questions stratégiques nationales

Nous avons tous été, nous sommes peut-être encore parfois et nous serons demain- si la loi scélérate sur le cumul des mandats est abrogée ! -des élus locaux. En tant que tels,

République : comme il n'est pas à l'île d'Elbe, il est inutile de demander le retour de l'Aigle- il fera ce qu'il souhaitera ! Ensuite, j'ai entendu beaucoup de choses : on nous explique qu'il faut qu'Engie reste une entreprise publique, parce que

mais pas pour un État propriétaire.

la stratégie de l'État en matière de production et de gestion du gaz naturel sur le territoire national. Je le redis, on constate un désengagement extrêmement fort d'Engie sur son coeur de métier

on constate- mais cela est passé assez inaperçu au cours des dernières années et le processus est encore en cours -une suppression et une externalisation, en Europe et à l'étranger, des centres de relation clients d'Engie.

; la seconde, c'est de penser essentiellement à l'échelle européenne. Car nous sommes des nains, avec tout le respect que j'ai pour nous-mêmes, par rapport aux colosses que sont les Chinois

Le scrutin est ouvert.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

La présence de l'État français dans le capital des entreprises n'a malheureusement pas d'effet sur leur comportement. Non seulement les entreprises dont l'État est actionnaire donnent la priorité au versement de dividendes, mais elles sont également parmi les plus actives en matière d'évitement fiscal. Ainsi Engie, dont l'État est actionnaire à hauteur de 24 %, possède 2 300 filiales, dont 327 sont basées dans des paradis fiscaux 133 aux Pays-Bas, 74 en Belgique et 28 au Luxembourg, où 27 milliards d'actifs ont été transférés et où Engie a même installé sa maison mère. Outre Engie, la Belgique attire entre autres EDF et Orange grâce à ces intérêts

qui m'ont demandé de vous poser une question, monsieur le ministre : trouvez-vous normal que les deux administrateurs de l'État qui siègent au conseil d'administration votent chaque année les schémas

Les réseaux électriques intelligents doivent constituer un levier essentiel de la transition écologique, et il nous semble que nous allons un peu vite en besogne sur le sujet. Nous regrettons que ce déploiement du nouveau réseau intelligent prototype se fasse sans concertation, à aucun moment, avec les usagers. Concrètement, le texte vise à faciliter les démarches pour les fournisseurs sans jamais demander leur avis aux usagers, aux « clients » comme on dit aujourd'hui. Il ne me semble pas très sage de faire comme si les craintes sur ce type de réseau n'existaient pas. En ce domaine, comme en d'autres, c'est bien le principe de précaution qui devrait prévaloir. L'exemple le plus connu- chacun le sait, car nous sommes régulièrement interpellés dans nos quartiers et nos localités -est celui du compteur Linky, qui donne lieu à de nombreux débats

les câbles accueillant la technologie CPL- courants porteurs en ligne -des compteurs ne sont pas adaptés aux 75 kilohertz. Bien évidemment, on ne peut attribuer tous les maux du monde au compteur Linky, puisque l'exposition domestique aux ondes vient tout autant des systèmes wifi, des téléphones portables et des télécommandes. Pour autant, l'effet cumulatif devrait, selon nous, être pris en compte. De fait, à défaut de pouvoir rassurer pleinement, le plus sage serait encore de faire preuve de patience, de travail et surtout de concertation en associant les utilisateurs aux expérimentations, de manière à n'avoir affaire qu'à des cobayes volontaires. Quel

les dérogations qui seront mises en place obéissent à un cadre strict et qu'elles seront notamment suivies de près par la Commission de régulation de l'énergie, laquelle devra à la fois les superviser et en assurer l'évaluation.

de l'État dans les conseils d'administration veillent au respect des règles fiscales par les entreprises. Je ne peux pas laisser dire que des administrateurs de l'État

Il n'est pas dans l'intérêt général que les grandes entreprises qui ont leur activité en France jouent au maximum l'optimisation fiscale contre le fisc. On pourrait à tout le moins espérer que les représentants de l'État attirent l'attention de ces grandes entreprises, dont vous nous dites qu'elles vont garder un certain sens de l'intérêt national. Permettez-moi d'en douter quand je vois leur manière de concevoir leur contribution à l'impôt

Il est toujours question des compteurs Linky. Mes collègues ont évoqué les inquiétudes d'un certain nombre de nos concitoyens au regard des risques pour la santé et les garanties à prendre. Ici, il s'agit plutôt d'être vigilant sur la question des données personnelles.

Sur le consentement exprès du consommateur, il est exigé pour l'enregistrement et la collecte de données plus détaillées, ainsi que pour la transmission à des tiers.

à habiliter la Commission de régulation de l'énergie ou les services de l'État à accorder des dérogations aux conditions d'accès et à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l'article L. 100-1 du code de l'énergie. Il est donc opportun que ces nouvelles dispositions ne soient pas mises oeuvre en totale méconnaissance de celles qui sont déjà prévues

à proposer aux gestionnaires des réseaux publics de distribution situés dans leur périmètre la réalisation d'un service public local de flexibilité portant sur des portions de ce réseau, afin de concourir à l'atteinte des mêmes objectifs de la politique énergétique. Par ailleurs, il est prévu que les dérogations puissent porter sur les articles L. 22-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, qui définissent les missions respectives dont sont chargés les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz dans leurs zones de desserte exclusives, conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies. En conséquence, il est essentiel que les autorités organisatrices susvisées soient directement associées aux dérogations ainsi accordées à titre expérimental par les services de l'État ou par la Commission de régulation de l'énergie,

de coordination. Il est essentiel que les autorités organisatrices puissent contrôler l'impact des dérogations accordées à titre expérimental par les services de l'État

Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement a pour objet de faciliter la mobilité réglementée, particulièrement des comptes d'épargne. En effet, en dépit de la mise en place de la mobilité réglementée, le taux d'attrition bancaire demeure très bas. Il est même en recul sur un an, passant de 4,8 % à 4,5 %, selon la Banque de France. L'un des freins majeurs à la mobilité réside dans la difficulté de transfert des comptes d'épargne, notamment réglementée, car un client ne peut détenir qu'un seul compte- livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d'épargne populaire, compte d'épargne logement, plan d'épargne logement et livret jeune-dans une seule banque. actuelle, ces livrets ne sont pas inclus dans le dispositif de mobilité réglementée, contraignant ainsi de nombreux clients à une potentielle multibancarisation non souhaitée et coûteuse. En effet, des frais bancaires sont également prélevés sur des comptes inactifs.

La clôture d'un livret d'épargne réglementée est gratuite, et l'ouverture d'un nouveau livret, immédiate. La concentration de la mobilité sur le seul compte courant représente plus un gage d'efficacité qu'une source de complexité.

Je n'énumérerai pas la longue liste des entreprises qui, quelque temps après leur privatisation ou la cession des actifs de l'État, se sont fait absorber

Ce mécanisme fait l'objet d'une rhétorique volontiers moderniste, puisqu'il doit marquer la fin d'une gestion « en bon père de famille [des] actifs de l'État dans un certain nombre d'entreprises », au profit d'un soutien à « l'innovation de rupture ». Cela sonne bien ! Ce soutien serait assuré par les intérêts tirés de la dotation initiale en numéraire du fonds, à hauteur de 10 milliards d'euros.

Conformément au principe d'universalité budgétaire, ce soutien peut être opéré directement par crédits budgétaires. Il peut également l'être par un fléchage des dividendes tirés des participations financières de l'État. Dès lors, si la nécessité de préparer notre pays aux évolutions futures ne semble guère devoir faire l'objet de débats, les modalités du soutien méritent d'être soigneusement examinées par notre assemblée. Je rappelle l'origine ancienne du projet de fonds pour l'innovation. Il trouve sa genèse dans la proposition d'un responsable de programme confronté à l'érosion progressive de sa dotation budgétaire. En effet, le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la banque publique d'investissement Bpifrance publié en septembre 2015 indique que, afin « de soutenir l'effort global de la Bpi en faveur de l'innovation, cette dernière a présenté un projet visant à instaurer une fondation dont la dotation budgétaire reposerait sur les dividendes assis sur un portefeuille d'actions actuellement détenues par l'Agence des participations de l'État. Ce système alternatif aurait pour but de compenser la baisse constatée de la dotation budgétaire du programme 192 et ainsi de permettre à la Bpi de verser davantage d'aides individuelles. » si les membres de la mission d'information comprennent la démarche de Bpifrance et partagent son inquiétude relative à la baisse de la dotation budgétaire, ils n'adhèrent cependant pas à la création d'une fondation dont le fonctionnement, tel qu'il est actuellement envisagé, conduirait à institutionnaliser un mécanisme un mécanisme de débudgétisation qui n'apparaît conforme ni aux règles de la loi organique relative aux lois de finances ni aux principes de vote et de contrôle du Parlement sur l'ensemble du budget.

Ce fonds est déjà créé et bénéficie d'une dotation hybride. Afin de prendre en compte l'action du fonds permise par le droit existant, il convient de maintenir l'article dans sa rédaction actuelle.

seront placés au Trésor, à un taux fixe de 2,5 % garantissant la stabilité de la rémunération sur les années à venir,

Aujourd'hui, Bpifrance n'est pas en mesure de toucher les produits de ces placements dans le compte du Trésor. Elle ne serait donc pas en mesure de dégager des moyens financiers pour investir dans les programmes d'innovation retenus par le Conseil de l'innovation.

précédemment, le fonds est déjà actif depuis un an et dispose de plus de 200 millions d'euros, pour soutenir, au titre de 2018, l'innovation. Il n'est pas avéré qu'une cession rapide des participations de l'État dans différentes entreprises s'impose pour financer l'innovation. D'autres solutions existent, comme en atteste la dotation actuelle du fonds. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

De par sa fonction et les intentions affichées à l'origine, Bpifrance devait disposer d'un fort ancrage local, matérialisé par la représentation dans ses instances dirigeantes des collectivités territoriales, à chaque échelon de la décentralisation propre à notre pays.

cette disposition n'est que le corollaire de la création du Fonds pour l'innovation et l'industrie opérée par voie réglementaire voilà un an. Ce fonds dispose d'ores et déjà des moyens de soutenir l'innovation, sans qu'il soit besoin de recourir au mécanisme financier proposé par le Gouvernement. Selon moi, il est donc logique de procéder à l'actualisation du Conseil d'administration de Bpifrance.

Bpifrance est depuis sa création adossée à la détention d'un certain nombre de titres et de parts d'entreprises publiques. Démonstration nous en est faite, d'ailleurs, par le fait que 13,3 % du capital d'EDF ont été cantonnés dans le bilan de Bpifrance pour assurer la mise en marche de la pompe à finance du Fonds pour l'innovation. On est, cela dit, assez loin de l'usage que nos voisins allemands firent, après la Seconde Guerre mondiale, de l'argent du plan Marshall, qui vint alimenter la célèbre la, établissement financier public qui, par une politique de prêts à faible taux d'intérêt, permit à l'Allemagne de conduire sa reconstruction et de conjurer l'un des maux endémiques de son économie, à savoir l'inflation. Aujourd'hui, dans un contexte où les taux d'intérêt sont faibles, notamment pour l'équipement des entreprises, nous aurions mieux fait de renforcer légèrement la centralisation de l'épargne populaire, par exemple autour du fameux livret A, pour proposer aux entreprises des prêts

présent amendement tend à assurer la compatibilité des actions de Bpifrance avec celles des réseaux consulaires, afin d'éviter la création de nouveaux services qui pourraient créer des doublons avec les actions déjà mises en place par ces établissements publics.

Depuis que ce texte est à l'étude, les dirigeants de notre pays essaient de nous dire que La Poste restera une entreprise publique. Il est vrai- c'est à noter -que la rédaction proposée conforte le caractère de service public de ses activités, maintient une exigence de détention publique et salariée du capital

De même, la nomination du président-directeur général continuera de relever de l'État et la présence d'un représentant de l'État au conseil de surveillance de la Banque postale est confortée. Mais le le changement de statut de l'exploitant public et sa soumission au droit commun des sociétés s'inscrivent dans un contexte de désengagement de l'État- personne ne peut le nier -et d'ouverture à la concurrence du secteur postal, désengagement et ouverture déjà largement engagés en vertu de politiques communautaires que que vous avez expressément soutenues en votant, au sein du conseil des ministres européen, la dernière directive postale. Forte de ces tendances, la direction de l'entreprise n'a eu de cesse de réduire les coûts pour réaliser des bénéfices au détriment des usagers et des personnels. Si nous ne pouvons soulever la question de l'inconstitutionnalité de toutes les décisions qui ont mis à mal le service public postal, nous allons faire la démonstration que ce projet de loi tend

! Plus sérieusement, je rappelle que cet article doit permettre à la société La Poste de renforcer ses activités notamment dans le domaine de l'assurance, un rapprochement avec CNP Assurances. Je veux surtout tordre le cou à toute crainte, peur ou fausse idée : en aucun cas cet article ne modifie les missions de service public de La Poste. D'ailleurs, il maintient la contrainte

du contrat d'objectifs et de moyens de La Poste, auquel je participe et auquel participent l'ensemble des organisations syndicales, a mis en évidence que, dès lors que le principe de l'actionnariat public est bien validé, ces dernières soutiennent toutes ce projet.

Le contrôle général économique et financier sera présent au sein de l'établissement et un commissaire du Gouvernement vérifiera le bon accomplissement par La Poste des missions de service public qui lui sont confiées par l'État. La composition du conseil d'administration sera aménagée, la représentation actuelle des salariés, à hauteur d'un tiers des administrateurs, étant conservée. Le rapporteur propose un poste de censeur supplémentaire afin d'assurer une représentation des élus locaux, et donc de la vision

que le volume du courrier a baissé de moitié en quelques années. De 7 % par an ! Les efforts de présence postale doivent donc forcément prendre une autre dimension. Heureusement qu'un grand nombre de collègues élus locaux comprennent cette nécessité et jouent un rôle de partenariat qui est précieux ! Mais dites-vous simplement que, si l'on n'avait pas développé La Banque postale et, maintenant, opéré le rapprochement avec la CNP, c'est-à-dire fait de La Poste un outil d'abord financier, il serait impossible de maintenir le niveau de présence postale que nous avons aujourd'hui et dont nous devons nous réjouir.

Nous avons besoin de continuer cette évolution, qui est exemplaire, de La Poste. Les techniques de communication ont profondément évolué

de La Poste, qui ont su évoluer. Alain Richard a eu raison de rappeler que le volume du courrier baissait. Nous communiquons tous par mail, et la communication écrite n'est en général qu'une confirmation de la communication numérique. Mais La Poste a su épouser la

Nous assistons aujourd'hui à ce miracle invraisemblable de la coopération entre le capitalisme international le plus agressif- je pense à la société Amazon -et la distribution des paquets. La Poste retrouve un nouvel élan. C'est elle qui porte à domicile ces millions de mètres cubes de cartons

la moderniser et lui donner toutes ses chances. Aujourd'hui, ce qui est proposé est en effet un sacrifice de la Caisse des dépôts et consignations, puisque la CNP devient un partenaire de La Poste. Réjouissons-nous d'avoir pour une fois

l'Observatoire national de la présence postale, que j'ai le plaisir de présider, met en place un contrat de présence postale territoriale, un budget de 174 millions d'euros, pour accompagner les collectivités. Ce sont ces dernières qui participent, les comités départementaux, à la présence postale dans le cadre de la mission d'aménagement du territoire de La Poste.

permettra au groupe de prendre une autre dimension et de transformer profondément son modèle économique. Pour mettre en oeuvre une telle transformation, le projet de loi prévoit de rendre l'État actionnaire minoritaire

L'actionnaire majoritaire sera à l'avenir la Caisse des dépôts et consignations, et non plus l'État. Si l'objectif affiché est de permettre une synergie- je dis bien une « synergie » -entre les 17 000 points de contact de La Poste et la force de frappe financière de CNP, il paraît essentiel de confirmer le principe de présence territoriale assurée par La Poste. Compte tenu de sa mission d'aménagement du territoire, La Poste dispose d'un maillage extrêmement précieux et d'un réseau de partenaires locaux tant publics que privés. Conformément à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 l'État, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité et La Poste s'engagent, dans le cadre de conventions adaptées et renouvelées, pour assurer cette présence territoriale. Au-delà de ses activités historiques, et le réseau des maisons de services au public, les MSAP, La Poste demeure l'un des derniers interlocuteurs de service public de proximité. Par cet amendement, nous souhaitons réaffirmer la volonté du législateur de maintenir cette présence postale territoriale et son adaptation aux besoins diversifiés des territoires et des populations, en développant non seulement ses services, mais également ses structures sur les territoires.

Je vous assure qu'il va y avoir un changement de nature avec ce qui va se passer. Les activités qui seront en place demain avec la CNP peuvent nous amener à faire des choix. Je préfère donc que le Sénat vote sur cet amendement.

par l'État et par La Poste indirectement.

est immuable ! Sur la question de la présence et des participations différenciées entre les territoires ruraux et urbains, je nous invite à avoir une analyse un peu plus fine et précise. Évidemment, La Poste ferme des bureaux en ville, ce qui pose aussi des problèmes. Évidemment, elle impose quand elle le peut des participations aux communes, y compris urbaines,

du service, en gardant la philosophie d'une péréquation pour garantir que les entreprises de service public et l'État travaillent de concert pour répondre à cette exigence. Sinon, nous ne parviendrons pas à rompre la logique infernale de l'accroissement des inégalités, dans laquelle on demande aux collectivités locales, pour éviter d'être complètement marginalisées, de financer des services que d'autres peuvent se payer parce que le marché, la solvabilité, la proximité le leur permettent.

les élus locaux étaient fort démunis. Le problème a commencé à être traité à l'échelle de la direction générale et de l'État, qui a la tutelle de l'entreprise,

En mai 2017, la Commission européenne a publié un document de réflexion économique faisant valoir que l'Union européenne ne doit pas être naïve dans son approche de la mondialisation. Les investissements étrangers représentent un enjeu fondamental. Ils façonnent le monde de demain et donc nos modes de vie. ces dernières années, les investissements directs étrangers, et plus particulièrement chinois, ont connu une progression spectaculaire. Ces investissements étrangers peuvent constituer parfois un risque majeur pour notre souveraineté. En renforçant l'arsenal juridique français comme le fait la loi PACTE, je pense que nous pourrons nous opposer avec plus de vigueur à la stratégie de pays qui agissent en véritables prédateurs pour prendre le contrôle de certaines de nos pépites.

Je soutiens donc cette démarche du Gouvernement prolongeant l'impulsion donnée à l'origine par Dominique de Villepin en 2005 et approfondie par le décret Montebourg en 2014. Cependant, je voudrais attirer l'attention du Gouvernement et de mes collègues. C'est bien de voter des textes de protection, c'est très bien de publier ensuite des décrets d'application, mais c'est encore mieux de les appliquer ! En cinq ans, le décret Montebourg n'a jamais été actionné ... J'espère que le texte qui sera voté aujourd'hui démontrera son utilité, surtout par sa mise en oeuvre. Je suis saisi de

: La parole est à M. Claude Kern. Cet amendement vise à clarifier l'article L. 151-3 du code monétaire et financier. Cet article prévoit que soient soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique relevant notamment de l'un des domaines suivants : activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale. Avec cet amendement n° 363 rectifié, nous clarifions la liste des domaines concernés et unifions la motivation du régime de dérogation à la liberté d'investir des investisseurs étrangers en France. Ainsi, seront soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l'ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire. Plus explicite, la présente rédaction s'applique à mieux appréhender les différentes composantes de la sécurité intérieure- ordre et sécurité publics -, comme de la sécurité extérieure- défense nationale tout en respectant nos engagements européens au regard des dérogations admises au principe de libre circulation des capitaux. La rédaction du présent amendement est de nature à garantir une meilleure prise en compte des enjeux spécifiques liés en particulier à la sécurité énergétique et alimentaire des Français. Sans nous soustraire à l'économie mondialisée, nous devons être en mesure d'avoir des garde-fous, car il y a des enjeux considérables en termes d'indépendance économique que nous devons préserver. Nous sommes plusieurs parlementaires sensibilisés à cette question, à laquelle j'associe naturellement l'ensemble des cosignataires de cet amendement, ainsi que mon collègue Olivier Henno.

Cet amendement étend la protection de l'État au foncier agricole, qui est le support de l'agriculture. Ces dernières années, les acquisitions de foncier agricole par des sociétés financières étrangères se sont accentuées. Pour trouver des mesures en vue d'endiguer ce phénomène, une mission parlementaire a été créée en 2018. Cependant, les achats massifs se poursuivent et nécessitent une réponse.

L'accaparement des terres en France est un vrai problème. Auparavant, aucune terre agricole n'était exploitée ou détenue par des sociétés. Aujourd'hui, 20 % des terres agricoles sont détenues par des sociétés. Il y a péril pour le mode d'agriculture familiale, mais aussi pour la sécurité alimentaire du pays.

d'investissements étrangers dans le foncier agricole, d'élevage ou viticole, dont les motivations à long terme ne sont pas toujours claires. Est-ce pour une production exportable, pour une production continentale ou européenne ? Cela reste à définir. À terme, ces investissements représentent un risque de perte de souveraineté dans le domaine alimentaire, alors que la sécurité de l'approvisionnement apparaît comme une nécessité, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Plusieurs initiatives ont été prises au niveau législatif et le décret du 14 mai 2014, dit Montebourg, a renforcé le dispositif réglementaire. Toutefois, cela reste encore insuffisant dans le domaine agricole. De même, les dispositions existant dans le code rural et de la pêche maritime visant à resserrer la maîtrise du foncier, en particulier le droit de préemption des SAFER, ne répondent pas totalement à l'objectif de cet amendement. C'est pourquoi il est proposé, dans le cadre de l'examen de ce projet de loi, d'inscrire les activités de nature à porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire dans le champ des activités soumises à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie,

La détermination des secteurs précis relève du décret, comme l'approvisionnement énergétique, l'approvisionnement en eau et la santé publique, qui sont déjà inclus dans le champ de ce contrôle.

le dispositif Montebourg est régulièrement utilisé chaque année, pour plus de dossiers qu'on ne le croit, et donne lieu à des décisions du Gouvernement. Je ne voudrais

pays d'Asie, et plus précisément la Chine, achètent des dizaines de milliers d'hectares en Afrique, mais aussi en France. Donc, sans avoir la

Mme la secrétaire d'État. Cet amendement vise à permettre à l'administration chargée du contrôle des investissements étrangers en France de requérir auprès des investisseurs étrangers toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, l'objectif étant d'améliorer les outils dont dispose le Gouvernement pour protéger nos entreprises sensibles et précisément instruire ces nombreux dossiers. À cette À cette fin, le texte que le Sénat a adopté en commission prévoit un renforcement significatif des mesures d'urgence, des mesures de police et des sanctions que le Gouvernement pourra prendre s'il constate des manquements. De manière prévisible, dans le contexte d'un contrôle plus exigeant, les décisions de l'État seront davantage susceptibles d'être contestées en justice. Les relations avec les investisseurs fautifs seront probablement moins collaboratives que lorsqu'il s'agissait de leur délivrer une autorisation pour investir. Cet amendement a ainsi pour objectif d'autoriser la direction du Trésor à requérir toutes les informations nécessaires pour exercer ses missions, à la fois pour instruire les décisions d'autorisation ou de refus, mais également pour démontrer le non-respect des conditions fixées. En effet, dans les décisions que nous prenons, nous pouvons poser des conditions, les les autorisations sous conditions étant ensuite étudiées au sein des comités de suivi. Il permettra de prévenir les situations dans lesquelles des investisseurs seront tentés d'invoquer le secret professionnel, le secret des affaires, pour ne pas remettre à l'administration les informations permettant de prouver leurs manquements.

Si son objectif est de mieux protéger les entreprises françaises sensibles, évidemment, nous y sommes favorables. La commission spéciale s'interroge toutefois sur la portée de cette obligation. C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat

n° 143. La constitution d'une délégation parlementaire serait la bienvenue pour renforcer le pouvoir de contrôle du Gouvernement sur un sujet aussi stratégique pour le pays que celui de la sécurité économique, liée également à la nature

issu d'une idée de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle, qui vise à répondre à la demande des députés d'être davantage associés au contrôle des investisseurs étrangers en France. Cet article a été adopté à l'unanimité des groupes politiques à l'Assemblée nationale- je me permets d'insister

une certaine importance aux usages -de créer une délégation commune entre deux assemblées sans concertation préalable et au moyen d'un amendement déposé sur un texte déjà en navette.

Je précise d'ailleurs que la commission spéciale a maintenu aux articles que nous venons d'adopter le principe de transmission par le Gouvernement aux assemblées des informations relatives à la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers.

à ce sujet. Il revient à chacune des assemblées d'organiser le traitement des informations comme elle l'entend, ce qui peut aussi passer par le biais du règlement.

sommes donc dans la continuité des échanges que nous venons d'avoir sur la sécurité économique et les investissements étrangers. Le Gouvernement est particulièrement vigilant à la sécurité et à la résilience des réseaux de communications fixes et mobiles et aux équipements qui constituent le coeur de ces réseaux. Avec le développement de la 5G qui est prévu dès le début de l'année 2020, les réseaux mobiles deviennent de plus en plus critiques du fait d'usages potentiels dans les domaines de l'industrie ou de la santé. Je vous donne un exemple

de l'importance de l'ensemble des enjeux actuels de sécurité nationale, notamment les risques potentiels de sabotage des réseaux. Cet amendement tend donc à soumettre à autorisation préalable du Premier ministre l'exploitation d'équipements actifs des antennes mobiles pour les opérateurs télécoms qui sont considérés comme des opérateurs d'importance vitale, dits OIV. Il a fait l'objet d'un avis positif de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, et a été élaboré avec les opérateurs télécoms concernés.

Ces mesures ne ciblent pas un équipementier en particulier. Des vulnérabilités peuvent être constatées chez tous les équipementiers et il convient de mettre en place les contrôles appropriés. La création d'un nouvel instrument juridique opposable pour contrôler les équipements télécoms n'emporte pas pas non plus un changement de doctrine de la France en la matière. Nous créons simplement les leviers nécessaires pour contrôler efficacement les équipements de réseaux et nous nous donnons la capacité de faire évoluer nos modalités d'action en fonction des évolutions technologiques. Il est évident que nous

Il est essentiel que ce nouveau régime n'obère pas la capacité des opérateurs à investir. Il leur faut un cadre juridique clair et transparent qui soit mis en oeuvre rapidement. L'amendement donne deux garanties très précises à ce stade : les autorisations préalables sont les plus larges possible, tant du point de vue matériel que temporel ou géographique ; les opérateurs connaîtront la liste des appareils et logiciels qui feront l'objet d'un contrôle. Le Gouvernement est évidemment prêt à poursuivre les travaux et, si nécessaire, à faire évoluer certains éléments du dispositif dans le cadre des travaux de la commission mixte paritaire.

L'absence d'adoption d'un tel amendement par la Haute Assemblée aurait des conséquences pour le moins paradoxales. D'une part, cela retarderait l'entrée en vigueur d'un dispositif qui me paraît essentiel par rapport à vos préoccupations de sécurité nationale.

Je m'étonne aussi qu'aucune étude d'impact n'ait été diligentée afin de mesurer les effets de cette proposition sur les investissements à venir, comme sur les matériels déjà installés. De plus, dans son avis du 4 février dernier, l'ARCEP relève l'ARCEP relève que la mesure proposée répond à l'objectif légitime de protection, de fiabilité, de sécurité et d'intégrité des réseaux de communications électroniques. Mais n'étant pas en mesure d'évaluer les risques encourus, l'Autorité se limite dans son avis à l'analyse des modalités de mise en oeuvre de la mesure proposée importera, en conséquence, dans la mise en oeuvre de ce dispositif, d'une part, que les modalités soient les plus claires possible et, d'autre part, que les effets rétroactifs, même indirects, soient évalués.

Bruno Le Maire a évoqué plusieurs points, sur lesquels je voudrais revenir. En premier lieu, il a exprimé son respect du travail parlementaire. Alors, acceptez que le Parlement ait le temps de mener les travaux nécessaires pour prendre les bonnes décisions

d'autant que, si les intentions du Gouvernement, que nous pouvons partager, pour renforcer la sécurité des systèmes d'information doivent être soutenues, un certain nombre de questions se posent. Je ne reviens pas sur l'absence d'étude d'impact. En outre, l'Europe semble s'être emparée de ce dossier. Mais quelle est sa position ? Quelles sont les orientations et les échéances d'une éventuelle évolution de ce dossier à l'échelle européenne ?

dans ce domaine et tente de faire quelque chose. J'ai bien compris que vous aviez envie d'avancer, puisque vous avez parlé de revenir en commission mixte paritaire pour faire encore évoluer votre proposition. Pour être très honnête, c'est la première fois, depuis que je suis élu, que j'entends dire que le Gouvernement dépose un amendement d'appel.

par les entreprises du CAC40, dont 57 milliards sont retournés aux actionnaires. Seuls 5 % ont bénéficié aux salariés

Rien sur la limitation des rémunérations des hauts dirigeants. Rien sur les avantages exorbitants qui leur sont consentis en dehors de leur rémunération principale. Et même, contrairement à vos déclarations qui laissent entendre que vous vous intéressez aux salariés, vous nous proposez des régressions.

le travail ». Si nous partageons ces objectifs, nous ne voyons pas leur concrétisation dans ce texte. C'est pourquoi le groupe CRCE avait déposé toute une série d'amendements qui s'inscrivaient parfaitement dans cette optique de justice et de partage. Nous avions déposé des amendements visant à partager les richesses créées. : l'un soumettait à cotisation les revenus financiers des entreprises, un autre revenait sur la transformation du CICE en allégement de cotisations sociales, un suivant réévaluait le SMIC et l'ouverture de négociations dans chaque branche professionnelle pour augmenter les salaires. Nous avions également déposé des amendements permettant de favoriser le dialogue social et l'intervention des salariés dans la gestion des entreprises. amendement accordant un droit de veto suspensif pour les représentants du personnel, à celui qui donne au comité d'entreprise un pouvoir de décision et de contre-proposition effectif ou à celui qui accorde des heures de délégation aux syndicats consacrées à l'information des salariés. déposé des amendements visant à mieux associer les entreprises aux problématiques sociétales : par exemple, le partage du travail par une réduction de la durée du travail à 32 heures par semaine, la responsabilité des entreprises à l'égard des salariés avec la suppression du barème des indemnités prud'homales ou encore l'interdiction des licenciements boursiers. Tous ces amendements ont été déclarés irrecevables. Alors que nos concitoyens réclament depuis des semaines plus de démocratie, alors que le Gouvernement prétend vouloir donner la parole au peuple dans le cadre de son grand débat national, le débat parlementaire, lui, est bridé. Le droit d'amendement se limite à une réaction au projet gouvernemental, tandis que toutes nos propositions qui répondent aux aspirations de démocratie et de justice sociale et fiscale sont rejetées.

... Cet article 57 me permet d'attirer votre attention sur le développement de l'épargne salariale, en particulier l'intéressement, dans le tissu des PME. Une amélioration et une extension du champ d'application de l'intéressement peuvent constituer pour de nombreux salariés une réponse à leurs attentes en termes de meilleure répartition des richesses et de progression du pouvoir d'achat. en 2016, seulement 17 % des salariés des entreprises de moins de 50 salariés étaient couverts par un dispositif de participation, d'intéressement ou d'épargne salariale et 11,1 % bénéficiaient d'un versement effectif. La même année, moins de 10 % des entreprises de 10 à 49 salariés avaient conclu un contrat d'intéressement ; ce sont surtout les entreprises qui se rapprochent de 50 salariés qui mettent en place ces contrats. Si, depuis dix ans, le montant distribué progresse légèrement- il n'est pas négligeable, puisqu'il représente 17 milliards d'euros en 2016 -, le nombre d'entreprises concernées et de salariés bénéficiaires a tendance à stagner. Le Gouvernement entend bien encourager les dispositifs d'épargne salariale, de participation et d'intéressement, en supprimant le forfait social sur l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés et sur la participation dans celles de moins de 50 Ces mesures vont avoir un effet positif immédiat pour les entreprises qui ont déjà mis en place des dispositifs sur la base du volontariat. Dans un deuxième temps, les salariés de ces entreprises devraient bénéficier de la suppression de ce forfait, car la plupart des entreprises raisonnent en fonction d'une enveloppe globale comprenant l'intéressement lui-même et les charges qui y étaient affectées. Mais cette mesure est-elle de nature à convaincre les entreprises d'opter, toujours sur la base du volontariat, pour ces dispositifs ?

ait donc un caractère obligatoire, avec des modalités qui pourront être encadrées par décret et négociées au niveau de la branche et de l'entreprise. C'est le sens de l'amendement que je proposerai à la suite de cet article. La parole est à M. Martin Lévrier, sur l'article.

C'est en effet un chapitre qui libère, en renforçant le lien employeur-salarié. Il supprime le forfait social versé au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur l'ensemble des versements d'épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il gèle l'intéressement au-delà d'un plafond au bénéfice de ceux qui sont en dessous. Il développe l'épargne salariale, ainsi que l'actionnariat salarié, et crée dans la loi une « société à mission L'article 1835 du code civil sera modifié pour permettre aux entreprises qui le souhaitent de se doter d'une raison d'être dans leurs statuts. Ce chapitre a pour vocation d'améliorer la transparence des sociétés cotées en matière de rémunération de leurs dirigeants au regard de la rémunération moyenne et médiane. Ce ratio d'équité contribuera à une responsabilisation accrue des pratiques salariales des entreprises. En outre, il sera, n'en doutons pas, un outil essentiel lors des négociations annuelles obligatoires. C'est aussi un chapitre qui donne une nouvelle visibilité citoyenne à l'entreprise. il modifie l'article 1833 du code civil pour consacrer la notion d'intérêt social de l'entreprise et la nécessité de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. également d'améliorer la parité femmes-hommes dans les directions des entreprises et de créer un label pour les entreprises qui mènent une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées. il instaure le fonds de pérennité, grâce auquel la France se dote d'un statut permettant de protéger de manière durable le capital de nos entreprises, pour assurer leur croissance à long terme. En réunissant toutes ces compétences, ce chapitre donne un nouveau souffle aux entreprises, ce qui leur permettra d'innover, de créer et de se développer. Ce texte rappelle à quel point l'épanouissement des salariés conditionne la réussite d'une entreprise. Pour illustrer ses intentions, rappelons-nous la citation du philosophe Jean Bodin : « Il n'est de richesse que d'hommes.

est à Mme Laurence Cohen. Cet article 57 s'inscrit dans le droit fil des articles dont nous débattons depuis la semaine dernière. Il intègre les modifications de seuils de l'article 6 et prolonge l'article 20, dont l'ambition était de réduire comme une de chagrin le montant du forfait social. Cet article supprime en effet le forfait social dans les entreprises de moins de 50 salariés, et il exonère les entreprises entre 50 et 249 salariés pour les versements liés à l'intéressement et à la participation. La commission des affaires sociales du Sénat a même été plus loin que le projet initial, puisque, pour les entreprises qui restent assujetties au forfait social, elle a abaissé le taux de 16 % à 10 %. Ces suppressions et diminutions du forfait social ont pour but de favoriser le recours aux dispositifs d'épargne salariale. Il faut rappeler ici que cette épargne n'a pas vocation à se substituer au salaire,

aussi une nouvelle niche sociale. Cette suppression appauvrit nos systèmes d'assurance chômage et retraite, qui sont pourtant des garanties essentielles permettant de sécuriser les salariés face aux aléas de la vie et de vivre mieux leur retraite. D'ailleurs, c'est, entre autres raisons, parce qu'il n'y a pas de cotisations sociales sur l'intéressement et la participation que le forfait social a été instauré. En supprimant ou en abaissant cette contribution, le Gouvernement prive la sécurité sociale de quasiment 700 millions d'euros, madame la secrétaire d'État. Cette mesure s'ajoute aux près de 50 milliards d'euros d'exonérations de cotisations sociales votées lors du PLFSS pour 2019, que notre groupe, évidemment, n'avait pas soutenues. Nous ne pouvons pas valider cette tendance. C'est pourquoi nous demandons avec force la suppression de cet article.

S'il est primordial de rééquilibrer le partage des bénéfices entre l'investissement, les actionnaires, et les salariés, il ne faut pas perdre de vue que l'essentiel du partage de la valeur ajoutée se joue en amont. Les bénéfices sont en effet la somme restante après que tous les autres postes de dépenses ont été pourvus. La maximisation des bénéfices est donc susceptible de se faire aux dépens de la part qui revient aux salariés dans l'entreprise sous forme de salaires, mais aussi chez les fournisseurs ou sous-traitants. En d'autres termes, une augmentation de la part des bénéfices attribuée aux salariés au titre de l'intéressement et de la participation peut être le fruit d'une série de choix en amont qui leur sont en réalité très défavorables- stagnation des salaires, licenciements, sous-investissement dans l'entreprise, etc. -, de même qu'à la collectivité dans son ensemble- répartition inéquitable le long de la chaîne de valeur, minoration de l'impôt, Réciproquement, mieux rémunérer le travail des fournisseurs, sous-traitants et salariés permet d'assurer un partage plus équitable de la valeur ajoutée en amont en faveur de ceux qui produisent en premier lieu les richesses de l'entreprise. De plus, les mécanismes d'intéressement et de participation utilisés pour associer les salariés à la réussite d'une entreprise s'accompagnent d'un risque majeur : celui de servir d'outil de flexibilisation des salaires, pouvant entraîner à terme une modération salariale et le report du risque vers les salariés. D'autres caractéristiques sont problématiques : ils bénéficient d'exonérations fiscales et sociales, sont dirigés vers des fonds de pension déconnectés de l'économie réelle, bénéficient principalement aux salariés des grandes entreprises déjà bien rémunérés, Loin d'être la panacée, les mécanismes d'intéressement et de participation ne doivent en aucun cas se substituer au salaire brut, sur lesquels employeurs et salariés versent des cotisations sociales et des impôts qui forment le socle du modèle français de solidarité et contribuent à réduire les

vous avez des comparaisons un peu rapides. Si je vous dis que 95 % des gens meurent au lit, cela ne fait pas du lit un endroit dangereux. Vous comparez

Allemagne, etc. Monsieur le rapporteur, nous avons l'habitude d'être presque en accord, même si nous ne partageons pas forcément les mêmes options, mais lorsque vous dites que, demain, tous les salariés vont pouvoir bénéficier de l'intéressement, vous allez un peu vite en besogne. c'est non pas une obligation, mais juste une incitation. En réalité, madame la secrétaire d'État, vous aviez trois possibilités pour faire en sorte qu'il y ait davantage de salariés qui puissent bénéficier des fruits de la croissance à l'intérieur de l'entreprise.

Je veux simplement faire un rappel historique. Le forfait social, à l'origine de l'intéressement- j'ai eu l'occasion de le pratiquer depuis plusieurs décennies -, c'était zéro.

CRCE que la ligne non pas éditoriale, mais politique d'Oxfam correspond à une certaine orientation. Elle est alimentée par un certain nombre de considérations, dont toutes ne sont pas nécessairement erronées. Effectivement, on peut considérer que l'intéressement, dans les entreprises qui le versent régulièrement, fait partie de la rémunération : il y a le salaire, qui est fixe et défini par des conventions collectives ou des accords de branche, puis l'intéressement, qui correspond à un partage des bénéfices.

Ce débat sur l'intéressement aurait pris une tout autre tournure si nous n'étions pas dans une période où le niveau salarial moyen dans ce pays n'était pas si détérioré,

de constater que, culturellement, c'est devenu un substitut à la hausse des salaires. Quand, en plus, on trouve un prétexte pour réduire les capacités de la sécurité sociale, qui, je vous le rappelle, est déjà rabotée par le Gouvernement,

C'est la preuve que nous consolidons financièrement notre sécurité sociale. Vous me parlez restrictions, mais quel gouvernement a mis en place le reste à charge zéro sur les prothèses auditives, sur les prothèses dentaires et sur les lunettes

Le scrutin est ouvert.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

%. Ce faisant, il augmente de 8 % à 10 % le taux de forfait social applicable aux sommes affectées à la réserve de participation pour les sociétés coopératives de production, les SCOP, tout en conservant le taux de 8 pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance. Cette hausse vient fragiliser l'équilibre économique des SCOP et diminuer la participation des salariés. Le présent amendement vise à conserver le taux actuellement applicable aux SCOP, actuellement applicable aux SCOP, dont la finalité est d'assurer le contrôle de l'entreprise par leurs salariés. Celles-ci bénéficient d'une gouvernance démocratique et d'une répartition des résultats prioritairement affectés à la pérennité des emplois et du projet d'entreprise. Pour ce faire, les résultats des entreprises sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives et aux salariés la participation à hauteur d'au moins 25 % des résultats, les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas. Dans une SCOP, les salariés détiennent au minimum 51 % du capital et des droits de vote. Leurs statuts peuvent d'ailleurs prévoir l'obligation pour les salariés d'entrer au capital de leur entreprise afin de participer à sa gouvernance. En vue de favoriser le versement aux salariés des résultats de leur entreprise, le code de la sécurité sociale prévoit un taux de 8 % pour le versement affecté à la réserve de participation. Une hausse du forfait social serait en contradiction avec la volonté actuelle de privilégier un modèle d'entreprise plus responsable,

terribles ! Le fait de traiter également des situations inégales ne va faire que renforcer les inégalités. C'est le danger qui nous guette,

vous allez pénaliser toute une série de coopératives, notamment celles de plus de 50 salariés. Elles ont impérativement besoin des 800 000 euros que vous allez ponctionner

pour la Nation, elle déstabiliserait cette voie très spécifique de bon partage des valeurs que constituent les sociétés coopératives de production.

participation. Le taux dérogatoire serait de 10 % pour toutes les autres, puisque le Gouvernement institue un taux dérogatoire à 10 % pour les abondements. Cela permettrait

qui est parfaitement louable, mais je crains que cette proposition n'induise de la complexité. Elle ne me semble donc pas souhaitable pour le moment. Il faut vraiment que le maximum d'entreprises s'engage dans ces dispositifs d'intéressement et de participation.

rectifié, parce qu'il vise à élargir le dispositif de suppression de taux de forfait social aux entreprises de 250 à 5 000 salariés.

est d'amener les entreprises à négocier rapidement des accords d'intéressement plutôt que de faciliter des accords qui existeraient sans cette incitation fiscale.

dit en même temps que l'économie sociale et solidaire, à défaut de constituer la matrice unique, concourt à une évolution positive en redonnant du sens au travail, en redistribuant de façon beaucoup plus saine la valeur,

Le scrutin est ouvert.